L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense

est favorable à l'adoption de ce texte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerce pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne

Quel est l'avis de la commission

amendement vise à préciser que, en cas de décès, d'incapacité ou de retraite d'un commerçant titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l'ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son son droit de présentation d'un successeur au maire en cas de cession du fonds de commerce. Le manque de précision du deuxième alinéa de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, combiné à des usages de terrain, laisse place à une interprétation extensive et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre les commerçants. Afin de mettre fin à des situations à l'évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l'ancienneté de l'autorisation d'occupation du titulaire initial ne peut être transmise à l'acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l'activité par son conjoint.

sens tend à préciser que, en cas de décès, d'incapacité ou de retraite d'un commerçant titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l'ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation

ou un marché et cède son fonds à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur.

du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l'amiable un titre d'occupation d'une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

doit se faire selon une procédure de sélection impartiale et transparente et selon des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Par ailleurs, il est déjà possible d'y déroger dans certains cas précis, par exemple s'il n'existe qu'un seul candidat ou si une première procédure de sélection s'est avérée infructueuse. Enfin, rien ne justifie d'exclure les halles et marchés de ce cadre, conçu pour garantir à tous les commerçants les mêmes opportunités. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Avec l'article 13 , nous poursuivons l'examen de la section 2 du chapitre I du projet de loi, laquelle section vise, aux termes de son intitulé, à simplifier la croissance des entreprises. Dans le cadre de nos travaux sur cette section, nous avions logiquement déposé plusieurs amendements concernant l'accès des PME à la commande publique. La commission spéciale a déclaré ces amendements irrecevables, considérant qu'il s'agissait de cavaliers. Elle estime donc que l'accès à la commande publique pour les PME n'a pas de lien direct ou indirect avec le projet de loi.

J'ajoute, au cas où ces éléments ne suffiraient pas, que le projet de loi, dans son article 63 , modifie le code de la commande publique. L'intitulé du projet de loi, ses chapitres et leur contenu attestent que l'accès des PME à la commande publique a toute sa place dans ce projet de loi. Les irrecevabilités prononcées par la commission spéciale ne constituent ni plus ni moins, selon nous, qu'un détournement de la Constitution. Constitution. Je reformule donc ma question, madame la présidente de la commission spéciale : au regard des règles constitutionnelles, en quoi ces amendements étaient-ils dépourvus de lien avec le projet de loi ?

si nous supprimions les CEPP, nous serions pris en flagrant délit d'instabilité législative. Tout en demandant le retrait de l'amendement, je remercie ses auteurs de permettre au Sénat de rappeler au Gouvernement ses vives

nous proposions dans une démarche constructive, afin de faciliter le rebond et de préserver l'emploi, d'instaurer un crédit d'impôt pour les établissements de crédit accordant, dans la limite de 100 000 euros, des prêts sans intérêts aux repreneurs individuels ou collectifs. Pour mesurer les données du problème, on rappellera ici que l'entreprise moyenne concernée par une transmission est en général une PME de 10 à 20 salariés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et dont le fonds de commerce est évalué à environ 800 000 euros. Autant dire que nous attendions de notre dispositif qu'il ait un puissant effet de levier et qu'il permette effectivement le dénouement de certaines reprises, préservant ainsi l'emploi et les activités économiques.

L'enjeu de soutien psychologique aux entrepreneurs dont l'entreprise connaît des difficultés nous paraissait pleinement répondre au contenu de cette section. Soutenir un entrepreneur en difficulté revient en effet à favoriser des possibilités de rebond. La décision d'irrecevabilité de notre amendement, au titre de l'article 45 de la Constitution, est donc incompréhensible pour notre groupe. Je vous demande

en procédure de redressement judiciaire est fixée par le juge-commissaire. Le projet de loi prévoit d'inverser le principe du droit en vigueur en maintenant la rémunération au niveau antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire. Pour notre part, nous considérons que le juge a d'ores et déjà les moyens de maintenir la rémunération des dirigeants en fonction de la taille de l'entreprise. La révision systématique du salaire du patron ne nous paraît pas indispensable, d'autant d'autant qu'une rémunération qui ne met pas en péril le redressement de l'entreprise peut être maintenue sans difficulté. En revanche, comment peut-on accepter des licenciements de salariés si les dirigeants touchent des rémunérations colossales représentant des centaines, des milliers, voire des millions d'euros ? Dans les petites entreprises, la rémunération du dirigeant peut représenter un montant important par rapport aux sommes en jeu. en jeu. Il est donc nécessaire de se poser la question de sa baisse, sans que celle-ci soit automatique. Nous sommes étonnés de constater que, d'un côté, le Gouvernement impose aux juges prud'homaux un barème des indemnités prud'homales et que, de l'autre, il supprime les critères légaux sur lesquels le juge-commissaire se prononce, car ils seraient « excessifs et incompatibles » et potentiellement susceptibles L'étude d'impact du projet de loi proposait de limiter l'automaticité du maintien des rémunérations des dirigeants en excluant les rémunérations manifestement excessives ou celles qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs visés par la procédure. Nous regrettons que cette option n'ait pas été retenue par le Gouvernement. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 14. Quel La commission a approuvé cet article que vous souhaitez supprimer, tout en simplifiant le dispositif proposé. Il s'agit de prévoir le maintien de la rémunération du chef d'entreprise en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire. Cet amendement étant contraire à la position de la commission,

une entreprise en redressement judiciaire, qui doit faire des efforts pour essayer de retrouver l'équilibre et repartir du bon pied, doit mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions possibles pour que cela puisse se réaliser. Je trouve donc

est rédigé, cet amendement ne concernerait pas les entreprises en redressement judiciaire, et il n'y a que 500 procédures de sauvegarde par an environ. de sauvegarde, l'administrateur judiciaire assiste généralement le chef d'entreprise dans sa gestion, sans avoir de rôle formel d'autorisation de ses actes. Le code de commerce précise en outre que, dans cette procédure, le chef d'entreprise peut accomplir les actes de disposition et d'administration de l'entreprise,

mais, dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées. Dans le cadre de l'élaboration d'un plan, les créanciers font régulièrement traîner la période d'observation en refusant d'adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S'ils agissent de cette manière, c'est qu'ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant, ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers, qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties. Il s'agit là d'une pratique préjudiciable à l'économie, puisque certaines structures sont liquidées, alors qu'elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits. Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n'agissent pas abusivement, loin de là. C'est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l'adoption d'un plan de sauvegarde. À ce titre, ils devraient se justifier par des motifs légitimes. On peut entendre par « motifs légitimes » le besoin d'avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n'est pas nuisible par rapport au débiteur. En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d'un créancier mal intentionné.

l'abus serait « sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de toute autre pénalité s'il n'est pas motivé par un motif légitime. ? Lors de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit consulter les créanciers sur les propositions envisagées pour régler leurs créances dans le cadre du projet de plan. Les créanciers peuvent accepter ou non ces propositions. Le plan est opposable à tous les créanciers. Pour les créanciers qui n'ont pas accepté ces propositions, le tribunal doit fixer dans le plan des délais uniformes de paiement. Dans ces conditions, tels qu'ils sont rédigés, les amendements n'ont pas vraiment de portée pratique, car ils visent un refus des créanciers lors de leur consultation sur les propositions de règlement envisagées dans le projet de plan. Dans cette hypothèse, la notion de refus abusif n'a pas réellement de sens d'un point de vue juridique.

Le fondement du droit des contrats est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives le consentement dans l'adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan, qui leur permet en quelque sorte de recouvrer leur créance à l'issue de Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire : en pratique, de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c'est proposer une solution ; ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate.

Il est défendu. Quel est l'avis de la commission spéciale ? Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous. Le plan s'impose donc aux créanciers, dans toutes ses dispositions. De manière générale, en cas de difficulté dans l'exécution du plan ou de l'accord, le chef d'entreprise doit saisir le tribunal, qui statue sur le problème. Tels que ces amendements sont rédigés, on ne voit pas exactement à quelle situation ils font référence.

le chef d'entreprise doit saisir le tribunal, qui statue sur le problème. Là encore, on ne voit pas exactement à quelle situation ces amendements font référence. En application du plan ou de l'accord, des remises de dettes ou des délais de paiement sont prévus. Dans ces conditions, comment les créanciers peuvent-ils ne pas respecter le plan,

Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiable de créances, et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et n'entraîne donc pas de frais en cas d'échec. L'explication est que le barème légal fixant la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement. Pourtant, il serait possible dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le parquet, liste qui est déjà prévue à l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel oblige les professionnels à déposer une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal d'instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue, tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure. Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens. Lorsqu'il ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire chargé de superviser le bon déroulement de la procédure et de prendre la décision d'autoriser certains actes concernant l'entreprise. Il désigne également des professionnels réglementés. Faire appel à une société de recouvrement de créances serait un changement assez substantiel, alors que le droit des procédures collectives prévoit justement des professionnels dont c'est la mission. Outre le coût supplémentaire que cela représenterait pour l'entreprise, ces sociétés ne sont pas soumises à des règles déontologiques particulières. Élargir le marché des sociétés de recouvrement de créances en les introduisant dans le système assez encadré des procédures collectives nécessite un encadrement juridique et déontologique plus important, sur la base d'une étude d'impact approfondie des pratiques actuelles qui en montrerait la nécessité. Cela ne peut pas se faire sans réflexion d'ensemble sur les acteurs des procédures collectives.

présenté l'an dernier au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, il est aujourd'hui plus simple de pousser une entreprise à mourir par un dépôt de bilan plutôt que de la fermer proprement. J'avais proposé un système de « turbo-dissolution » inspiré de ce qui existe dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, qui faciliterait le rebond.

Je comprends parfaitement pourquoi le Sénat a voulu supprimer cette mention : pour éviter de stigmatiser le chef d'entreprise. Simplement, je pense que d'autres arguments plaident en faveur de ce rétablissement.

Deuxième argument : il s'agit de prévenir le cas où un chef d'entreprise pratique des liquidations judiciaires à répétition. Il nous paraît important que cela soit porté à la connaissance de ceux qui pourraient décider de reprendre l'entreprise. Il me semble essentiel

spéciale ? On ne peut pas, dans le même mouvement, vouloir favoriser le rebond des entrepreneurs de bonne foi qui ont rencontré des difficultés, y compris une liquidation judiciaire, et défendre la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire, comme si c'était une condamnation pour une infraction pénale. De plus, cette mention au casier judiciaire ne concerne que les entrepreneurs individuels, mais pas les dirigeants d'une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui crée une rupture d'égalité caractérisée. L'objet de l'amendement fait également état de la nécessité de vérifier l'absence de liquidation judiciaire en cours comme condition pour ouvrir une procédure de rétablissement professionnel : le projet de loi supprime justement cette condition. Enfin, le travail des parquets en matière commerciale peut s'appuyer sur les vraies sanctions, qui resteraient bien sûr mentionnées au casier et qui concernent les entrepreneurs malhonnêtes ou particulièrement incompétents, y compris les dirigeants de société et pas seulement les entrepreneurs individuels. L'avis est donc défavorable.

qui touchent l'ensemble des organismes de sécurité sociale -, la mention paraît nécessaire. De toute façon, les magistrats savent très bien que si l'entreprise est de bonne foi, cette mention ne figurera pas au casier ou, en tous les cas, peut en être radiée. donc très hésitante sur la suppression de cette mention du casier judiciaire.

telle mention au casier judiciaire implique qu'on assimile une liquidation judiciaire à une infraction. Or la liquidation judiciaire, c'est la constatation

possible par ce biais. Sanctionner par une inscription au casier judiciaire des liquidations simples de personnes de bonne foi est une peine supplémentaire pour ceux qui cherchent à faire face à leurs

telle que l'obtention d'un plan de redressement judiciaire. Elles ne sont pas des sanctions à l'encontre de l'entrepreneur ayant connu l'échec et ne reflètent en aucun cas la capacité de gestion de ce dernier. Il s'agit de marqueurs objectifs appelant les établissements de crédit à faire preuve de vigilance. En réalité, ces cotations sont très handicapantes. Les établissements de crédit, plutôt que de prêter attention, rejetteront purement et simplement toute demande de financement de l'entrepreneur faisant l'objet d'une cotation 050 ou 060, et ce alors même que le juge a considéré que l'entreprise était encore viable et que c'est particulièrement à ce moment qu'un soutien financier serait nécessaire au rebond de l'entrepreneur.

C'est ce que nous voulons supprimer.

La liquidation judiciaire entraîne un certain nombre de droits qui peuvent être parfois assez importants. Je pense principalement à l'AGS, le régime de garantie des créances des salariés : n'importe quelle personne en France peut créer une société fictive, embaucher une dizaine de personnes de sa famille ou des prête-noms,

libellé : La parole est à Mme Jocelyne Guidez. Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois, les textes régissant les sanctions en la matière n'évoluent pas au même rythme. S'agissant de la liquidation judiciaire, il n'apparaît pas opportun que la personne physique n'ayant pas encore fait l'objet d'une sanction professionnelle, comme la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, voie inscrit à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité. Cette inscription a pour effet de mettre à l'index toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire, alors même que l'ouverture de celle-ci peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même.

est à Mme Sylvie Vermeillet. Le privilège de prêteur de deniers permet au prêteur d'être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier : si celui-ci doit être saisi et vendu, le prêteur titulaire de ce privilège peut être indemnisé en priorité. Actuellement, le privilège de prêteur de deniers est souvent préféré à l'hypothèque conventionnelle, car c'est une garantie moins coûteuse pour l'emprunteur, n'étant pas soumis à la taxe de publicité foncière. Or l'article 16 du projet de loi, sous couvert de simplification, propose de supprimer le privilège de prêteur de deniers au profit du dispositif de l'hypothèque légale, alors que, pour le client, il peut y avoir un manque à gagner. Par exemple, le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros par rapport à un prêt avec privilège de prêteur de deniers. Pour ces raisons, il est proposé de conserver le privilège de prêteur de deniers, dans l'intérêt même des clients emprunteurs. Quel Quel est l'avis de la commission acheter en VEFA. Ce privilège n'est donc pas utilisable dans tous les cas, notamment pas pour des opérations mixtes. L'étude d'impact est néanmoins extrêmement succincte sur cette réforme, pourtant importante pour les particuliers comme pour les entreprises

pour l'administration fiscale que pour les entreprises, l'étude d'impact évoque un relèvement du seuil d'inscription de 15 000 à 200 000 euros par décret. Il s'agit d'un élément aussi important, voire davantage, que ce qui est prévu dans le projet de loi lui-même, car les conséquences de l'inscription peuvent être

Un outil existe pour informer les salariés dans toute entreprise : la banque de données économiques et sociales, définie par l'article L. 2312-36 du code du travail.

figurent certains dispositifs et informations qui peuvent toujours s'avérer utiles pour le comité social et économique de l'entreprise. Toutefois, il manque des données essentielles en matière de fiscalité.

Notre dernier amendement reprenait une proposition d'une commission d'enquête du Sénat, présidée par notre collègue Philippe Dominati, qui préconisait de créer un délit d'incitation à la fraude fiscale. Pourquoi avoir déposé ces amendements ? Tout simplement parce que la lutte contre la fraude fiscale est l'affaire de tous, ... Eh oui ! ... notamment des salariés, ne serait-ce qu'en raison de l'obligation de dénoncer tout fait délictueux. Par ailleurs, alors que l'on

amendement vise à remédier à certaines difficultés relatives à la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement à partir de laquelle s'apprécie la fin du semestre civil et en précisant que le montant au-delà duquel l'inscription doit être prise s'apprécie créance par créance à l'issue du semestre civil, et non de façon cumulée. Quel est l'avis du Gouvernement ? Avis favorable.

Si l'intention est bonne, il est en revanche regrettable de devoir constater que ce texte ne va pas toujours assez loin. Quand une entreprise connaît des difficultés, elle reste soumise à ses obligations fiscales. Pour l'accompagner, il existe divers mécanismes de report, d'aménagement, de conciliation.

Actuellement, la prise en considération des difficultés de l'entreprise relève majoritairement du pouvoir discrétionnaire de l'administration et du comptable public. Pour l'entrepreneur connaissant des difficultés, la sécurité juridique afférente à ces dispositifs est donc relativement faible, et le refus d'octroi d'un avantage qui lui semblait légitime peut mener à la mise en péril de son activité. Il y va pourtant de l'intérêt de l'entrepreneur comme de celui de l'administration fiscale : une entreprise qui dépose le bilan est une entreprise qui ne concourt plus à la bonne santé économique du pays ni à celle de ses finances publiques. C'est la raison pour laquelle, dans mon rapport d'information relatif à l'accompagnement du cycle de vie des entreprises, j'avais proposé de réviser les mécanismes de modulation des pénalités et majorations de retard, notamment en instaurant leur progressivité en lieu et place de la linéarité

%. La logique d'accompagnement des entreprises par les services collecteurs a déjà pu être enclenchée l'année dernière par l'instauration du droit à l'erreur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas l'avoir davantage développée à l'occasion de l'élaboration du présent projet de loi ?

de reprise. Ce dispositif, adossé à l'épargne salariale, permet au salarié d'utiliser l'argent dont il dispose sur le plan d'épargne d'entreprise pour abonder un fonds de reprise, lequel rachètera des parts de l'entreprise en question, faisant ainsi du salarié un actionnaire. Si l'idée à des salariés de participer à la reprise de leur entreprise est plutôt séduisante, la manière dont elle est mise en oeuvre ici est peu satisfaisante : ce dispositif n'est finalement rien d'autre que le parent pauvre des coopératives. En effet, bien souvent, les salariés sont actionnaires minoritaires, et n'ont pas de réelle possibilité de participer à la gestion et à la prise de décision dans l'entreprise.

ils ne détiennent que 16 % des parts de la possédant ces deux entreprises. Ainsi, les salariés, lorsqu'ils se regroupent, restent largement minoritaires, et de plus la voix des salariés considérés individuellement n'a aucun poids. En fin de compte, les salariés financent l'entreprise qui les emploie sans vraiment avoir leur mot à dire ; au mieux, ils ont la possibilité de participer au noyau dur des actionnaires stables. Pour avoir un réel poids et prétendre être majoritaires, ils devraient rassembler une somme considérable au regard de leurs revenus, surtout quand il s'agit de grandes entreprises dont les parts valent cher. D'ailleurs, ce dispositif est assez discriminant tous les salariés ne disposent pas d'une épargne, et tous ne peuvent pas épargner à la même hauteur. Ceux qui pourront acheter des parts en grand nombre sont ceux qui ont les revenus les plus importants.

parole est à Mme Laurence Cohen. L'article 19 supprime l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Cette obligation est issue de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, dite « loi Florange ». À l'époque, notre groupe avait regretté que le texte ne concerne que les grosses entreprises, de plus de 1 000 salariés, mais cette loi obligeait les groupes voulant fermer un site rentable à rechercher un repreneur pendant trois mois, ce qui était tout à fait positif.

Pour l'entrepreneur cédant, l'opération de reprise d'entreprise par les salariés représente la possibilité d'assurer une transmission en douceur et en confiance, avec des repreneurs qui connaissent déjà l'entreprise. Il y a moins de risques que l'opération soit abandonnée avant la signature ou que les données collectées pendant la transaction fuitent vers la concurrence, par exemple. Pour les clients, les avantages tiennent au fait d'avoir des interlocuteurs inchangés et très motivés, qu'ils voient progressivement monter en responsabilité. Si plusieurs salariés sont repreneurs et ont une vision solidaire de l'entrepreneuriat, avec des principes de gouvernance partagée, le recours à une société coopérative de production s'inscrira dans une démarche solidaire et responsable, que nous défendons par ailleurs. Je pense notamment aux anciens salariés de Fralib, qui ont créé la marque de thé « 1336 », que je vous recommande, mes chers collègues ! Quel est l'avis de la commission spéciale ? Restreindre le bénéfice de cette exemption de droits sociaux aux seuls salariés de l'entreprise paraît contestable dans son principe, et conduirait par ailleurs à la création d'une taxe supplémentaire. La commission spéciale

exiger l'attestation du paiement total de la prime dès le début de l'année conduirait les assureurs à revoir les conditions de souplesse accordées aux assurés pour échelonner les paiements. Il en va de même pour les attestations de chantier, puisque la prime définitive est calculée à la fin du chantier. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet alinéa. Quel est l'avis de la commission

dont certaines ont connu, notamment au cours des deux dernières années, la faillite, et ont laissé sans aucune couverture de nombreux particuliers et collectivités.

Cet amendement vise à compléter les modifications apportées par le projet de loi aux règles d'éligibilité des juges des tribunaux de commerce, définies par les articles L. 723-4 et L. 723-7 du code de commerce.

d'une possible défaillance, appelant des mesures préventives. La préoccupation ayant inspiré l'amendement adopté par la commission spéciale est satisfaite par d'autres dispositions de procédure assurant la communication d'informations utiles à la juridiction consulaire. Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du CODEFI, comme l'a souhaité l'Assemblée Quel est l'avis de la commission spéciale ? Les informations « signaux faibles » sont de nature à permettre d'anticiper les difficultés qui pourraient compromettre la continuité de l'exploitation, avec plus ou moins deux années d'avance. Leur transmission permet au président du tribunal de commerce d'assumer sa mission de détection des difficultés des entreprises le plus en amont possible. C'est la raison pour laquelle le tribunal de commerce doit bénéficier, en raison de ses compétences, des mêmes sources d'informations que les autres instances membres du CODEFI. La commission a donc émis défavorable sur cet amendement.

sur les sociétés et d'un accès au fichier national des interdits de gérer.

Les informations figurant dans ces fichiers ne lui seront donc d'aucune utilité pour exercer sa mission, qui ne concerne pas la prévention des difficultés des entreprises. Ainsi, ces amendements ne semblent pas vraiment répondre au problème qu'ils soulèvent. C'est la raison pour laquelle la

n° 72 rectifié. Lors de son arrivée à la tête de l'entreprise, le repreneur peut découvrir que certaines réglementations ou législations n'ont pas été scrupuleusement suivies. Ainsi, en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné. Une telle situation peut bloquer certaines transmissions. Par ailleurs, elle fait peser un risque inconsidéré sur les épaules du chef d'entreprise, qui n'est pas responsable de la situation et n'est pas à même de la régler dans l'instant.

et de leur application à toutes les entreprises sans distinction. Ils posent un problème au regard du principe constitutionnel d'égalité entre les entreprises, mais aussi entre les salariés d'entreprises différentes. Par ailleurs, les règles de protection des consommateurs ou de l'environnement pourraient-elles, en bloc, être ignorées pendant six mois ? Est-ce envisageable pour de graves atteintes à l'environnement ? Un commerçant alimentaire devrait-il pouvoir ignorer gravement les règles d'hygiène, sans pouvoir être sanctionné par la DGCCRF ? Les manquements ne pourraient pas être sanctionnés, qu'ils soient graves ou légers, volontaires ou non. Les infractions pénales seraient-elles concernées ou non ?

Toutefois, la retraite supplémentaire reste marginale au regard de l'attractivité des autres produits d'épargne. À titre de comparaison, l'encours de l'assurance vie

De plus, le montant des rentes d'épargne retraite reste relativement faible par rapport aux prestations versées par les régimes de retraite obligatoires.

à l'objectif du Gouvernement de dynamiser l'épargne retraite supplémentaire. Elle estime que la portabilité des droits, l'harmonisation des règles de fonctionnement des produits d'épargne retraite

Par conséquent, elle a adopté un amendement, sur l'initiative du rapporteur, fixant à 10 % le taux du forfait social sur ces versements. Ces quelques points du rapport au fond que je viens de rappeler montrent bien où l'on veut en venir. Finalement, peu de salariés ont commencé de participer aux plans d'épargne retraite existants, malgré les incitations diverses, notamment fiscales.

Cependant, elle ne finance pas assez la croissance des entreprises : seulement 11 % de l'épargne des Français est alloué au financement des fonds propres des entreprises,

Les fonds propres nets des sociétés non financières représentent en France 66 % du PIB, contre 123 % aux États-Unis et 52 % en moyenne dans la zone euro. Nous devons donc créer une structure de financement beaucoup plus orientée vers le renforcement

à être versée. Aucun autre choix n'est possible : pas de sortie en capital, uniquement une sortie en rente viagère ! Une telle orientation ne peut évidemment pas recevoir notre assentiment, car, au-delà de la méthode mise en oeuvre par le Gouvernement,

Il va sans dire qu'une telle démarche ne peut pas nous agréer. Il est indispensable que la sortie en capital soit autorisée, notamment pour tous les salariés qui, proches de la fin de leur carrière professionnelle, n'auront pu cotiser suffisamment longtemps pour constituer une épargne digne de ce nom.

des salariés à la vie de l'entreprise, afin qu'ils se sentent véritablement concernés par les résultats, les bénéfices, les progrès réalisés. Cela étant,

de la Fédération française de l'assurance en date du 30 mars 2017, 55 % des détenteurs d'un contrat âgés de 35 à 59 ans utilisent l'assurance vie pour préparer leur retraite. Une partie d'entre eux le font en plaçant leur épargne sur des fonds euro, qui offrent des rendements limités et obèrent la capacité des sociétés d'assurances à investir dans l'économie réelle. Cet amendement vise donc à permettre à celles et ceux qui le souhaiteront de transférer leur épargne des fonds euro vers un plan d'épargne retraite sans frottement fiscal.

La finance et l'économie sociale et solidaire, l'ESS, répondent à des logiques et à des règles différentes. Les marchés financiers sont cantonnés à certaines classes d'actifs. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne sont pas, pour l'immense majorité d'entre elles, des entreprises émettant des actions. Pour pouvoir investir dans les entreprises de l'ESS, les sociétés de gestion d'épargne salariale ont su, depuis vingt ans, innover et s'adapter. Ainsi, s'agissant de la part investie en actifs solidaires, 70 % des lignes d'investissement des

des titres éligibles à une liste fixée par voie réglementaire.

sécurisés. Quand on parle retraite, on parle aussi sécurité et garanties, quelle que soit la sortie, en rente ou non. En outre, la liste des titres pouvant être acquis dans le cadre de l'épargne retraite doit être fixée par voie réglementaire. Il faut simplement faire attention à ne pas donner trop de place au pouvoir réglementaire.

offrant une protection suffisante », dont la liste exhaustive doit être fixée par décret en Conseil d'État. J'espère que cette précision vous rassurera,

Ainsi, par ce mécanisme, une quote-part des placements pourrait être affectée aux zones où le PIB par habitant et/ou le seuil de pauvreté sont les plus bas. Un tel dispositif serait particulièrement pertinent s'agissant de zones comme la Guyane, où les besoins sont plus importants qu'ailleurs

les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l'obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l'offre de placement de l'épargne salariale, selon une proportion dite « 90-10

dans le cadre de la gestion pilotée. Je suppose qu'il s'agit d'un oubli. Après trois ans, la gestion pilotée concerne déjà 40 % des encours des PERCO,

dit, il faut une transparence totale. Je ne suis pas défavorable à ce que les épargnants puissent investir dans des fonds solidaires, mais je voudrais surtout que l'on évite la confusion entre gestion pilotée et investissement

il pourra désormais, grâce à l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, investir son épargne retraite dans des fonds solidaires. Un tel geste est utile pour l'économie sociale et solidaire, à laquelle je crois profondément, mais il faut être honnête avec l'épargnant

Je partage ce que vous avez dit, monsieur le ministre : placer son épargne dans l'économie sociale et solidaire est un acte militant, qui ne relève pas de la simple recherche du bénéfice maximum.

termes de votre amendement, c'est « dans le cadre d'une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers »- cela correspond très exactement à la définition de l'épargne pilotée -« qu'une partie des sommes recueillies [pourrait] être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires